chers collègues, afin de limiter la circulation de documents, vous êtes invités à utiliser vos tablettes et la fonctionnalité « En séance » sur notre site internet

Voilà un amendement qui devrait nous permettre, monsieur le rapporteur, de commencer ce débat dans une grande sérénité ... En effet, notre groupe propose de prévoir, s'agissant de la quarantaine et de l'isolement,

Êtes-vous prêt à le faire ? Si tel est le cas, la commission des lois suivra Mme Rossignol.

pendant la période de confinement. Je suis donc au regret de lui dire que je confirme l'avis favorable de la commission. Il est bon que, dans cette période particulière, des dispositions particulières s'appliquent en faveur des femmes et, plus rarement, des hommes victimes de violences conjugales.

raison -à mon administration et à tous ceux qui ont travaillé sur ce texte. Je ne voudrais surtout pas que l'on puisse conclure que je ne serais pas favorable à cette disposition,

Il nous paraît concevable qu'une personne, même contaminée et soucieuse de ne faire courir aucun risque à autrui, puisse, dans des conditions contraintes, bénéficier de possibilités de sortie compatibles avec le respect des gestes barrières.

à cette personne un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant d'échanger librement avec l'extérieur. Ces précautions sont évidemment Toutefois, qu'adviendra-t-il si ces conditions ne sont pas réunies ? Le présent amendement vise à prévoir que, en cas de non-respect de ces conditions, la mesure de placement en quarantaine ou à l'isolement sera nulle et non avenue. Quel est l'avis de la commission

soient mieux proportionnées aux circonstances de temps et de lieu. En effet, pour que ces mesures soient efficaces d'un point de vue sanitaire, il est nécessaire qu'elles permettent de réduire la densité afin de limiter au maximum les interactions entre individus. Beaucoup d'observateurs ont noté des incongruités, tel l'accroissement du nombre de personnes se promenant dans les centres de villes balnéaires parce que les plages étaient interdites. Parallèlement, dans les métropoles, il a pu paraître parfois contre-productif de réduire les plages horaires pour la pratique d'activités individuelles les lieux de circulation des personnes, ces mesures ayant pour effet d'accroître la densité dans les plages horaires et les lieux de passage permis. C'est pourquoi il est proposé de prendre en compte cette notion de densité. Cela se justifie totalement dans le cadre d'un état d'urgence destiné à lutter contre une épidémie. L'Aubrac, avec ses deux habitants au kilomètre carré, n'est pas comparable au front de mer de Biarritz et aux berges de la Seine ou du canal de l'Ourcq.

Il s'agit de ne pas se résigner, de réinventer des moyens de vivre nos libertés dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, tout en prenant les dispositions sanitaires nécessaires. Quel

commission ? Je remercie notre collègue Françoise Gatel et les cosignataires de cet amendement d'avoir soulevé cette question. Elle intéresse beaucoup de maires en France.

et les pouvoirs de police générale qui sont ceux des maires. Les pouvoirs de police générale des maires ne s'exercent que par exception quand un pouvoir de police spéciale est donné au préfet. Il ne faudrait pas créer un risque de compétition

nous ont réclamé de limiter les possibilités d'engagement de leur responsabilité à raison des décisions qui relèvent de leur compétence, et voilà que nous élargirions par la loi le champ de leur responsabilité, et donc celui des poursuites

monsieur le ministre,

Je suis élu de l'Oise ; ma collègue Laurence Rossignol pourra vous confirmer que l'on observe actuellement une épidémie d'arrêtés de fermeture ou de non-réouverture d'écoles dans notre département. Si l'on suit le raisonnement de notre cher président de la commission des lois, tous ces arrêtés sont illégaux- c'est ce qu'il nous a fait comprendre hier.

pour régler le problème posé par l'amendement de Françoise Gatel, serait plutôt que, dans un rapport de partenariat, le maire estimant n'être pas en capacité d'assurer soit les services périscolaires, soit la bonne organisation des locaux pendant le temps scolaire

fermer l'école ou, au contraire, de passer outre, considérant que les arguments ou les données de fait présentés par le maire sont insuffisamment probants. Je fais la distinction entre la mise en état des locaux, locaux, strictement indispensable au fonctionnement du service public scolaire, et la fourniture des services périscolaires, car ces derniers ne sont pas obligatoires.

la réalité vécue par nos collègues maires et par les directeurs d'école. Je m'empresse de dire, pour l'avoir moi-même vécu, comme la plupart d'entre vous j'en suis sûr, des échanges quasi hebdomadaires que nous avons avec les préfets et l'ensemble des représentants de l'État territorial, que ledit État territorial sollicite pleinement les maires. Je prendrai un exemple.

monsieur le ministre,

En ces temps de crise, le discernement dans la sanction de nos concitoyens et concitoyennes devrait être de mise. Comment justifier, par exemple, le fait de punir des femmes et des enfants lorsque ceux-ci violent les mesures d'urgence sanitaire afin d'échapper à des violences intrafamiliales, lesquelles sont en train d'exploser depuis le début du confinement ? Cette situation est d'autant plus problématique que les témoignages se multiplient, dévoilant les faits d'une verbalisation parfois irrégulière, abusive et ciblée, notamment dans certains quartiers populaires. Le nombre de contraventions dressées est ainsi trois fois plus élevé en Seine-Saint-Denis que sur le reste du territoire français, alors que nos banlieues connaissent actuellement, comme vous le savez, une détresse sanitaire, sociale et alimentaire grandissante. Il n'est vraiment pas nécessaire de les stigmatiser encore davantage. Enfin, mes chers collègues, le placement en garde à vue, la comparution immédiate et l'incarcération potentielle des personnes mises en cause risquent de créer un brassage problématique et inopportun en cette période de pandémie. Alors que les sanctions aux manquements à l'état d'urgence sanitaire devraient viser à contenir le virus, en l'occurrence, elles pourraient favoriser sa propagation.

du nouveau coronavirus, mais il peut en rester. Or je ne vois aucune raison de supprimer la possibilité d'appliquer les sanctions pénales, à savoir les amendes,

est à Mme Laurence Cohen. À l'heure actuelle, quelque 3,5 millions de propriétaires forestiers possèdent les 12,2 millions d'hectares de la forêt privée. D'après le cadastre, environ 380 000 propriétaires forestiers possèdent plus de 76 % de la surface forestière, de 4 hectares à plus de 100 hectares. Ces chiffres montrent que le poids des propriétaires forestiers privés ou particuliers est non négligeable, et que leur gestion responsable et durable est essentielle. L'article L. 112-2 du code forestier dispose en outre : « Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. « Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique. les incendies liés aux sécheresses accumulées ces dernières années sont de plus en plus récurrents et peuvent devenir incontrôlables. Dans un motif d'intérêt général de préservation des bois et forêts forêts et de leurs voisinages, alors que nous entrons dans la saison sèche, il est donc nécessaire de permettre aux propriétaires forestiers de limiter tous risques d'incendies dans leurs forêts et leurs bois. Les dispositions de la présente loi doivent donc autoriser les propriétaires particuliers à se déplacer, pour effectuer tous les travaux d'aménagements, tels que le débroussaillage,

je suis comme le parti communiste : je défends la propriété forestière et foncière. J'ai donc du mal à émettre un avis défavorable sur cet amendement, qui est inspiré par un excellent motif. Toutefois, je suis obligé de vous le dire, mes chers collègues, vous n'avez pas besoin de faire adopter cet amendement pour que les propriétaires forestiers puissent entretenir leurs parcelles et prévenir les incendies, qui sont à l'heure actuelle la principale cause de la précarité de leurs revenus. Vous avez

qui serait complété par un suivi dans le cadre d'un protocole conçu plus globalement et précisé dans l'objet de cet amendement, le tout placé sous le contrôle du préfet et de l'agence régionale de santé, l'ARS. Un second test est d'ailleurs prévu à J+3 ou J+5 dans le projet développé par la collectivité de Saint-Barthélemy.

Les avis défavorables- j'y faisais référence -de la commission et du Gouvernement reposent notamment sur l'absence de fiabilité des tests pour déterminer si une personne est assurément contaminée au moment où elle entre sur le territoire. Parallèlement, le dispositif prévu à l'article 2 prévoit la possibilité, pour le préfet, de prononcer une mesure individuelle de confinement, sur constatation médicale. Comment cette « constatation médicale » sera-t-elle obtenue, monsieur le ministre ? Faut-il considérer que les personnes arrivant de pays dans lesquels le virus a circulé devront être systématiquement soumises à un examen médical à l'arrivée ? En tout état de cause, cet examen ne comprendra-t-il pas un test ? On comprend bien que conditionner l'entrée sur les territoires ultramarins à une période de quarantaine revient à exclure toute reprise de l'activité touristique, dès lors, que concrètement, on obligerait tous les touristes à ajouter quatorze jours à leur période de vacances. ces territoires peuvent au contraire être « pilotes » de la réouverture de notre économie nationale. Il ne s'agit pas, en outre, d'ouvrir l'accès aux touristes dès le 11 mai, mais d'en créer les conditions en inscrivant dès à présent la base légale qui le permettra, le moment venu, en assurant la sécurité sanitaire. Quel enfants. Quel est l'avis de la commission ? Magras, coauteur de cet amendement. Il est vrai que les restrictions à l'entrée sur le territoire d'un certain nombre de collectivités d'outre-mer empêchent la reprise de l'activité touristique.

en l'efficacité du test de dépistage pour prévenir les risques de contamination, alors que celui-ci n'est pas infaillible. Quand le test révèle la contamination,

-d'extrapoler votre conclusion pour l'inviter dans le débat sur la carte des départements, représentés en vert ou en rouge. Si l'on admet que la fiabilité des tests doit être portée dans le débat public, pourquoi en avons-nous fait l'un des trois items qui permettent de déterminer la couleur des départements ? Il est important

est à M. le ministre. Madame la sénatrice, je n'ai pas de famille antillaise, mais c'est parce que j'aime profondément les Antilles que je ne prendrai pas, à titre individuel, la responsabilité de risquer de transmettre le virus là-bas.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, L'article 3 du présent projet de loi prévoit les modalités de placement à l'isolement des citoyens contagieux. Une telle décision serait prise par le représentant de l'État dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et après constatation médicale. Un garde-fou est prévu, le juge des libertés et de la détention, pouvant être saisi par le patient. Malheureusement, la rédaction présentée par le Gouvernement n'est pas vraiment satisfaisante. Rappelons-le, la mise à l'isolement pour raison médicale est une privation de liberté, alors même que le porteur du virus n'a rien commis d'illégal. Cette décision n'est donc pas à prendre à la légère et doit être encadrée. Le présent amendement tend donc à proposer une nouvelle rédaction de l'article 3, afin que le placement coercitif en quarantaine se dote d'un cadre légal rigoureux garantissant la nécessité et la proportionnalité d'un recours à une telle mesure. Le dispositif que nous proposons appelle notamment à se faire plus respectueux du droit à l'information et à la défense de la personne placée à l'isolement. Il y est notamment prévu la garantie de la présence d'un avocat dans le cadre de l'audience du malade avec le juge des libertés et de la détention. Il y est également assuré que le requérant se verra informé par écrit, et dans une langue qu'il comprend, de la nature, de la durée et des motifs de la mesure à laquelle il est soumis, ainsi que des droits qui lui sont reconnus. La rédaction proposée ici devrait permettre de concilier un dispositif proportionné et respectueux des droits des personnes concernées avec les moyens dont disposent les autorités pour agir contre la propagation de l'épidémie.

vise à préciser qu'une mise en quarantaine n'est possible que si l'infection est établie ou si la personne refuse de se soumettre à un test de dépistage ou à un examen médical. Pourquoi ? Parce que les conditions de mise en quarantaine et de mise à l'isolement, ainsi que la distinction entre ces deux catégories, ne sont pas suffisamment claires parce qu'aucune disposition n'a encore été prise aux frontières pour organiser ce qui constitue une mesure privative de liberté et parce qu'il nous semble que mieux vaut un dépistage qu'une quarantaine sans test préalable. Enfin, rappelons que, depuis la mi-mars, le Gouvernement a incité les Français installés à l'étranger à ne pas rentrer en France. De plus, l'organisation du rapatriement de plus de 150 000 personnes fut concentrée sur les personnes

Comment concilier des décisions individuelles et le droit de mener une vie familiale normale, droit protégé à l'échelon national et européen ? Il est certainement encore trop tôt pour évaluer les effets du confinement sur les enfants, lequel ne peut pas tout à fait être comparé à l'expérience d'un

afin de préciser que le juge statue par une ordonnance motivée pour garantir des conditions de recours satisfaisantes à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle de mise en quarantaine ou de placement

Monsieur le ministre, vous pouvez maintenir votre amendement, mais je suis obligé d'émettre un avis défavorable, car il est contraire à la position de la commission. Et je ne pense pas que cela ait une réelle importance

nous sommes devant un sujet d'importance d'un point de vue constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a, selon moi de façon extrêmement judicieuse, fixé cette séparation

doit être regardée comme privative de liberté une mesure qui entraîne l'impossibilité d'aller et venir plus de douze heures par jour. Lorsque je vous écoute décrire les modalités de ces mesures, certes d'ordre médical,

Nous voterons contre cet amendement si vous ne le retirez pas et nous serons favorables à l'amendement tendant à prévoir que l'ordonnance doit être motivée, quand bien même elle doit l'être en principe. La parole est à M. le ministre.

vise à mettre en place, comme chacun le sait, de nouvelles mesures d'isolement et de mise en quarantaine. Ce dispositif impose des mesures de privation de liberté très restrictives pour les personnes concernées. En effet, le placement à l'isolement ou la mise en quarantaine serait prononcé par le préfet, sur proposition de l'agence régionale de santé. Dans le dispositif proposé par le Gouvernement, aucun contrôle de cette privation de liberté

qui sera ainsi appelé à statuer dans les quarante-huit heures sur un placement en isolement décidé par le préfet. Je sais que cela peut apparaître contraignant, mais il s'agit, mes chers collègues, des libertés, et le Sénat, vous le savez, est très vétilleux- il a raison de l'être -sur ces questions.

Lors de la présentation de la stratégie nationale de déconfinement devant l'Assemblée nationale, le mardi 28 avril 2020, M. Édouard Philippe

« Notre politique repose, à cet égard, sur la responsabilité individuelle et la conscience que chacun doit avoir de ses devoirs à l'égard des autres. Nous prévoirons des dispositifs de contrôle, s'ils devaient être nécessaires, mais notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun. » Cet amendement vise à tirer les conséquences de cette déclaration, que nous jugeons particulièrement importante.

La quarantaine et l'isolement, par nature, sont des régimes de contrainte, ce qui n'est pas le cas, par nature, du système de prescription médicale, qui vous invitera à vous mettre en quatorzaine si vous avez approché un porteur du virus.

Comme le souligne son président, « le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi que dans le seul cas d'une privation absolue de la liberté », lorsque toute sortie est interdite, tandis qu'est supprimée toute possibilité de recours

argué que l'ouverture des écoles est essentielle pour les enfants en situation difficile,

Mesdames, messieurs, chers parents, « Dans le cadre du plan de déconfinement, le Gouvernement a annoncé la réouverture des écoles maternelles et primaires le 11 mai. « Pour la santé de nos enfants et du personnel enseignant, ce protocole est difficilement applicable, sachant que notre région est en zone rouge, que le conseil scientifique préconise une rentrée des élèves en septembre et que des cas graves chez les enfants apparaissent dans les hôpitaux limitrophes de notre département. Dans ces circonstances, sachant qu'un maire a un devoir de protéger sa population, j'ai pris ce jour la décision de maintenir la fermeture des écoles de notre commune au-delà du 11 mai, avec une réouverture

décrit la situation de fonctionnement de l'établissement scolaire, mais ne statue absolument pas sur l'hypothèse d'une fermeture et donc d'une réouverture.

trouve ici ses limites. Il faut toute la finesse du président de la commission des lois pour interpréter, en s'appuyant sur la jurisprudence, l'article L. 411-1,

qualifiées, susceptibles d'apporter une expertise technique au Gouvernement. Cela ne dispense pas le Gouvernement d'être en lien étroit avec les usagers

en continu se déroule hors du cadre du conseil scientifique, dont les missions sont de rendre des avis scientifiques

Le conseil scientifique a pris une place considérable dans notre vie publique. Par moments, il a donné l'impression

soit nommé dans des conditions plus transparentes et que le Parlement ait un rôle plus important à jouer

corriger des décisions que nous avons prises il y a peu de temps, dans la loi du 23 mars. Pour autant, les délais urgents dans lesquels nous travaillons ne nous permettent pas toujours d'être aussi excellents, performants et rapides que nous voudrions l'être.

alors que l'État français disposait en 2009 d'un stock de 723 millions de masques de protection FFP2, en mars dernier, seuls 80 millions de masques chirurgicaux étaient encore utilisables par nos services hospitaliers. Ces chiffres interpellent, mais n'étonnent guère lorsque l'on connaît les maux structurels de la France. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs se sont appliqués à démanteler notre service public de santé. Ce santé. Ce constat va de pair avec la réalité d'une France globalisée, qui a abandonné son indépendance sanitaire à des puissances étrangères comme la Chine. Bien que l'exécutif l'ait nié au début de la crise, il est désormais reconnu que le port du masque est essentiel à la non-propagation du virus. Vous vous êtes enfin décidé à le rendre obligatoire, par exemple dans les transports, ce qui est une excellente décision. Nous aurions pu saluer cette mesure si sa mise en oeuvre n'était pas la parfaite illustration de votre orientation libérale. Alors que vous auriez pu marquer le grand retour de l'État social par une politique industrielle publique ambitieuse, qui aurait permis de distribuer des masques à chacun, notamment aux plus précaires, vous avez fait le choix de laisser le secteur privé à la manoeuvre. Dans les jours à venir, 500 millions de masques inonderont- nous l'espérons ! -les grandes surfaces et les pharmacies. Où étaient ces masques quand nos soignants en avaient besoin ? Où sont désormais les mesures de plafonnement de leur prix, pour les rendre abordables pour tous ? Cette crise nous aura appris que le que le nouveau monde n'a de toute évidence rien appris des erreurs de l'ancien.

Ensuite, depuis le début de la crise, mon groupe est extrêmement critique sur les choix politiques qui sont faits en matière de santé par ce gouvernement, qui a amplifié les choix précédents et qui n'a pas l'air de tirer de leçons de la crise terrible que nous vivons. Monsieur le ministre, je ne doute ni

Monsieur le président, « J'ai procédé à une commande en Chine de masques FFP2 et de lunettes en date du 6 avril 2020, tous produits à la norme CE.

La commande est prête à être livrée de Chine sur la France, mais- c'est là le problème -le service des douanes de la cellule Covid-19 de Roissy-Charles-de-Gaulle multiplie les barrières administratives : traduction de tous les documents et, surtout, revalidation des masques par un laboratoire français. « Depuis le début de la pandémie, le CH- je ne le nomme pas -, établissement de santé mentale de troisième ligne, fonctionne sur des livraisons de dotations d'État en flux tendus depuis six semaines. Cette situation devient intolérable pour les médecins et les soignants, les agents hospitaliers et les gestionnaires, qui voient en vente libre des masques en grande distribution, quand, aujourd'hui, la pénurie de masques ne nous autorise pas à rouvrir des structures

monsieur le ministre. « Chères consoeurs, chers confrères, « Les masques FFP2 délivrés dans les pharmacies après accord entre le Conseil national de l'ordre et le ministère de la santé ne seront pas disponibles avant lundi, si tout va bien. Ce n'est pas de la mauvaise volonté des pharmaciens. Ils sont obligés d'attendre les instructions officielles de délivrance du ministère et les masques qu'ils ne recevront peut-être pas pour lundi. Dans l'attente, le conseil départemental est en mesure de distribuer quatre masques à chaque praticien en activité du département, dotation d'État livrée au Conseil. Vous pourrez venir les chercher à partir de ce mardi, de

de Lidl expliquer qu'il commandait des masques avec l'autorisation du Gouvernement depuis le mois de mars dernier. C'est normal, puisque les supermarchés sont ouverts et qu'il est absolument nécessaire que les patrons

que, pendant tout le mois d'avril, il manquait des masques pour les soignants. Vous comprendrez, monsieur le ministre, qu'il y a tout de même un sérieux problème de régulation de la part

Depuis peu, la production de masse a repris de façon très abondante en Chine. Comme nous avons été les premiers à passer des commandes nombreuses, nous avons été parmi les premiers. Je ne rappellerai pas les épisodes dignes d'un western sur les tarmacs des aéroports chinois,

Monsieur le ministre, je ne serais pas intervenu si vous ne nous aviez pas soumis cet argumentaire, qui est un justificatif de ce qui s'est passé avec les masques.

Le décret de réquisition apparaît comme un acte d'une force administrative extraordinaire. Il a eu pour effet d'assécher tous les circuits. L'État a été incapable de commander,

des mesures de confinement avaient entraîné le besoin d'une plus grande harmonisation dans la pratique de verbalisation sur le territoire national ici, on contrôlait le contenu d'un caddie ; là, on demandait un ticket de caisse ; ailleurs, on reprochait à quelqu'un d'être allé chercher son pain à bicyclette au lieu de l'avoir fait en voiture ... Tout cela est remonté à l'échelon national, et l'on s'est rendu compte qu'il était très difficile

des agents verbalisateurs des chemins de fer et de la RATP, qui sont rompus à l'exercice de dresser des procès-verbaux.

qu'arrive cette demande du Gouvernement de donner des pouvoirs dérogatoires au droit commun à des personnes qui ne sont pas formées pour les exercer. C'est la raison pour laquelle la commission des lois

il y aura une récupération vers une remise en ordre de marche des autres fonctions de la police et de la gendarmerie, ce qui justifie de trouver des renforts.

L'article 5 permet d'habiliter un certain nombre de personnels pour faire respecter les mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence, Philippe Bas vient d'en parler. parler. Il donne en particulier aux agents assermentés des transports publics la faculté de faire respecter l'obligation du port du masque, leur conférant des pouvoirs de police étendus relevant de l'ordre public, alors que les mesures de police traditionnellement exercées par ces agents relèvent le plus souvent de la sûreté et de la sécurité ferroviaires. Nous formulerons tout d'abord une remarque sur la forme. Il est incroyable que, à notre connaissance, les organisations syndicales du secteur, tant à la SNCF qu'à la RATP, n'aient pas été consultées sur de telles mesures.

ni souhaitable ni utile. C'est aux forces de l'ordre de faire respecter l'état d'urgence et les mesures y afférentes et non aux agents du service public, alors que l'habilitation est très large. Ainsi, ce sont plus de 17 000, voire 20 000 agents, qui pourraient se voir chargés de nouvelles missions. est d'autant plus important de le souligner que nous savons qu'il faudra mobiliser de nombreux agents pour faire respecter la distanciation dans les transports, si tant est que l'on y arrive, pour accueillir les voyageurs et, ce qui serait encore mieux, pour participer à la distribution de masques gratuits, comme cela se fait dans d'autres pays européens. Pour toutes ces raisons, il ne faut pas donner à ces agents des tâches supplémentaires de verbalisation des personnes qui ne porteraient pas de masque. Nous demandons donc la suppression de ces dispositions, en considérant que la seule mission incombant aux agents des transports publics doit être de renseigner, d'accompagner les usagers et de faire en sorte que la sécurité sanitaire soit assurée dans les transports, notamment en ce qui concerne le flux des voyageurs.

dispose, depuis une loi du 1 janvier 2014, que les membres des forces de l'ordre doivent porter sur leur uniforme un numéro d'identification. Cette obligation d'identification s'applique aussi aux personnels verbalisateurs dont le code des transports régit l'action.

et je ne sais toujours pas si est réglé, aujourd'hui, le problème concret qui va se poser quand plusieurs centaines de personnes arriveront, par exemple, à une bouche le métro,

et pour que l'on puisse retrouver dans la rame une personne tous les deux sièges, sans personne debout. Je ne sais pas si ce problème est réglé, monsieur le ministre, mais j'aimerais que vous nous apportiez des précisions sur le sujet, car je suis très inquiet de ce que nous a dit le Premier ministre, ou plutôt de ce qu'il ne nous a pas dit.

dresser procès-verbal en cas d'infraction aux règles posées pour l'urgence sanitaire. L'amendement du Gouvernement, à rétablir le texte initial, toujours sur cette question de la verbalisation. Nous n'y sommes pas favorables non plus. Enfin, je voudrais dire, à propos de l'amendement n° que chacun sait ici la haute idée que le président Sueur se fait de la fonction parlementaire et du rôle de la loi. Pour autant, je ne trouve pas que cet amendement soit tout à fait à la mesure de cette haute idée,

par l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure. Puis-je vous suggérer plutôt, monsieur Sueur, de demander au Gouvernement de prendre une circulaire Ce sera un moyen plus approprié pour rappeler une obligation réglementaire que l'inscription de ce rappel dans la loi. Si le Gouvernement veut bien

ainsi libellé : La parole est à Mme Esther Benbassa. L'article 5 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les agents agissant dans les transports publics et ferroviaires de verbaliser les usagers qui ne respecteraient pas les mesures sanitaires édictées à l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, en ne portant pas de masque. Nous comprenons évidemment l'objectif du Gouvernement visant à responsabiliser nos concitoyens par des mesures coercitives, afin d'éviter au maximum la transmission du Covid-19. Philosophiquement, une telle mesure est en revanche contestable. Les Français dans leur ensemble ne se comportent pas comme des mineurs et ils comprennent parfaitement le besoin de respecter les règles sanitaires édictées par l'État. Leur sens du civisme aurait probablement suffi. C'est une vision optimiste, mais l'heure n'est pas à la polémique, et nous saluons le choix du Gouvernement, qui semble tendre vers un port obligatoire du masque dans les transports en commun, comme le préconise l'ensemble de la communauté scientifique.

de la pénurie de masques que connaît notre pays depuis le début de l'épidémie, une mise en pratique de cette mesure ne soit pas possible dès le 11 mai. Il semble donc particulièrement injuste de pénaliser nos concitoyennes et concitoyens en les verbalisant pour non-respect des règles sanitaires, alors même que c'est l'État qui est le principal responsable du manque de masques. Le présent amendement vise à corriger cette injustice, en autorisant la verbalisation de nos concitoyens dans les transports uniquement si l'application des normes sanitaires est matériellement possible. C'est bien à l'État de réunir les conditions essentielles à la sécurité sanitaire de chacun, notamment en donnant la possibilité aux citoyens

réintroduire la possibilité pour les capitaines de navire de procéder à des contrôles, de manière à nous permettre de lutter efficacement contre la diffusion épidémique. Quel est l'avis de la commission ?

à des fins exclusives de pratique sportive de pleine nature. Dans le cadre du déconfinement progressif, il a été précisé que les activités sportives, dites « de pleine nature », seront de nouveau ouvertes aux pratiquants, au même titre que les autres activités sportives.

L'autorisation explicite de ces pratiques dans un cadre raisonné permettrait, mes chers collègues, non seulement la relance des activités économiques, mais aussi une démarche progressive- j'insiste sur ce terme -, d'appropriation du littoral en amont de la saison estivale. L'accès aux plages sera bien évidemment encadré par un protocole validé conjointement par le maire et par le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.

aux familles de retrouver une vie la plus normale possible, dans le respect de l'ensemble des gestes barrières, selon le vocable utilisé.

Il s'agit d'amendements qui visent en réalité la liberté de circulation, laquelle est restreinte, ou peut l'être, en application de l'état d'urgence sanitaire. À mon sens, si une interdiction générale et absolue d'accéder aux plages pouvait éventuellement se comprendre pendant la période du confinement, elle est beaucoup plus difficile à justifier en période de déconfinement. On peut se demander si la limitation au droit d'aller et venir ne serait pas disproportionnée par rapport aux fins visées, à savoir la sécurité sanitaire. Il y a des petites plages et des grandes plages ; il y a des plages à la ville et des plages à la campagne. Ainsi,

Les risques de contamination y sont maîtrisés, jusqu'à présent. Enfin, il y a aussi des plages où la position verticale est de mise, et celles où la position horizontale est privilégiée. Vous le voyez, dans cette diversité, appliquer un traitement unique a véritablement quelque chose de tout à fait excessif. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, il me semble qu'il serait prudent, du point de vue du respect de cette liberté fondamentale qu'est la liberté d'aller et venir, que le Gouvernement revoie sa position d'interdiction générale et absolue et permette d'inverser le principe, en prévoyant la liberté, sauf exception qui serait justifiée par l'impossibilité d'éviter la promiscuité sur les plages, que vous décideriez ainsi d'interdire au public pendant une durée limitée. est la recommandation que je voudrais vous faire. À cet égard, je considère que ces amendements sont l'un et l'autre extrêmement intéressants. Par conséquent, le Sénat pourrait fort bien les adopter.

l'on peut faire ou non respecter les gestes barrières et la distanciation physique sur les plages. Je suis convaincu, comme vous, qu'un maire totalement responsable, en collaboration avec un préfet, est fondé à prendre des mesures pour faire respecter

sommes tous intimement convaincus : si l'on rouvre les plages, l'activité touristique va repartir, ce qui sera formidable pour l'activité de notre pays, mais formidable aussi pour le virus.

Je m'aperçois, monsieur le président, que j'ai été incomplet. Il faut bien que je vous dise vers lequel de ces deux amendements pourrait aller notre préférence. Il me semble que l'amendement présenté par notre collègue bellilois de Haute-Savoie, M. Loïc Hervé, présente des avantages, compte tenu de ce que vient de dire le ministre. Comme cette disposition renvoie à un décret, elle permet au Gouvernement de déterminer les conditions dans lesquelles des décisions de fermeture temporaire pourraient être

je pense, identique. Je suis solidaire de la Bretagne, bien sûr, mais aussi de la Vendée dans cette revendication. En effet, si des parcs sont amenés à être rouverts, si l'accès à la forêt est de nouveau autorisé, les plages aussi méritent toute notre attention. L'avantage des plages du nord, c'est qu'elles bénéficient de marées. À marée basse, l'espace est encore plus large pour s'égailler et surtout pratiquer le confinement actif lorsque l'on fait du sport. Je soutiendrai cet excellent amendement, d'autant que notre président de région,

l'île d'Ouessant. Elle n'est pas très connue pour ses plages, mais elle est célèbre pour sa qualité de vie, l'art de vivre et la fierté de ses habitants de pouvoir aller voir leurs voisins

explication de vote. Monsieur le ministre, je suis prêt à vous entendre sur le fait qu'il faille encore attendre. Mais la patience pèse aujourd'hui sur l'état psychique

Je faisais le calcul dans ma tête : il y a à peu près 4 millions de personnes dans ma région qui se trouvent à moins de 100 kilomètres d'une plage. Donnez-leur un espoir de pouvoir retrouver une vie normale ! Je l'ai entendu tout à l'heure, le Président de la République aurait évoqué la date du 2 juin pour autoriser

fermement l'amendement qui a été présenté par mon collègue Loïc Hervé. J'espère que vous tiendrez compte de la forte

et je fais confiance au maire de Dinard ou de Saint-Malo, lesquels, avec le préfet et sur avis de l'ARS, donneront l'autorisation, dans un cadre extrêmement réglementé,

progressive du littoral feraient beaucoup de bien en cette première période de déconfinement.

Il n'est pas facile d'être législateur. Il y a les rats des champs et les rats des villes ; il y a les élus, cher Philippe Bas, des plages de la campagne et les élus des plages de la ville.

raison pour laquelle je suis très sensible au discours du président de la commission des affaires sociales. Le combat contre l'épidémie n'est pas terminé.

de l'incertitude où nous sommes encore sur la rapidité de circulation du virus. Comme ma collègue qui siège en face de moi, je fais des allers-retours entre les deux départements, Paris et le Val-d'Oise, où la circulation du virus est la plus forte.

Si nous faisons passer le message que la fréquentation des lieux de vacances que sont les plages, les forêts et les chemins de montagne est rouverte pour les locaux,

d'Alain Milon. Son statut de médecin lui confère une autorité que nous sommes peu nombreux à avoir ici. Néanmoins, si l'on va jusqu'au bout de sa logique, il ne faut pas déconfiner

se trouvent partout sur le territoire. Tout à l'heure, avec beaucoup de bon sens, Ladislas Poniatowski a dit que les gens ne comprenaient pas pourquoi on pouvait s'entasser dans un supermarché et ne pas aller dans une forêt où il y a une personne au kilomètre carré.

Si on déconfine, on s'intéresse non pas à des lieux, mais à des pratiques. Sur une plage, on peut être assis sur une serviette de bain, sans bouger, avec des enfants faisant des châteaux de sable à moins de 50 centimètres ; on peut aussi avoir des pratiques sportives qui sont totalement différentes. S'agissant des pratiques de pleine nature,

L'adhésion, la responsabilisation, la capacité des individus à prendre en considération pour eux-mêmes et pour les autres les règles sont tout aussi importantes que la force des règles qu'on leur impose. Selon moi, avec de telles précautions, on peut autoriser les pratiques de pleine nature, notamment sur les plages.

En effet, les premières victimes sont les personnels de santé, qui, notamment au début de cette crise sanitaire, manquaient parfois de matériel de protection. Surtout, au-delà même des risques que ces auteurs d'infraction font courir aux personnels de santé et à la population tout entière, les bénéfices financiers qu'ils peuvent susciter sont choquants et intolérables. intolérables. La presse a relaté à plusieurs reprises des cas de trafics illégaux. Certains ont même organisé du porte-à-porte pour revendre des masques, jusqu'à 15 euros l'unité ! Face

pour tout vol commis en période de menace ou de crise sanitaires grave, portant sur un bien de première nécessité destiné à prévenir ou à limiter cette crise ou cette menace. Les peines seraient ainsi portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

de nombreuses inquiétudes ressurgissent quant à l'accès aux tests pour les personnes, qu'il s'agisse de professionnels ou non, qui interviennent dans des lieux d'habitation. C'est le cas des aides à domicile, mais aussi des millions d'aidants qui oeuvrent quotidiennement auprès d'un proche malade, en situation de dépendance ou de handicap. Parce qu'elles participent à l'effort de la Nation, parce que certaines d'entre elles ont subi la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, parce que toute une chaîne de la solidarité nationale se serait dissoute sans leur mobilisation, ces personnes méritent l'attention des pouvoirs publics.

Entre les contraintes professionnelles et familiales, leur intervention n'est pas toujours facile en temps normal. En pareilles circonstances, elle l'est encore moins. À l'épuisement physique et psychologique, n'ajoutons pas une prise de risques

Nous devons être capables de tester tout le monde, de tracer tout le monde, d'isoler tout le monde et de casser les chaînes de contamination ; ainsi, nous serons sûrs que l'épidémie est redescendue à un niveau suffisamment bas pour être maîtrisée.

Monsieur le ministre,

La durée de validité des titres de séjour a été prolongée par le Gouvernement, parce que les services des préfectures, chargés de ces procédures, étaient largement à l'arrêt. Néanmoins, à partir du 11 mai, le travail reprendra.

le tribunal administratif de Paris s'est prononcé très récemment- à la mi-avril -pour ordonner non pas que l'on ferme le centre de rétention administrative, mais

rationnels conduisent à fermer les centres de rétention administrative pendant le temps, finalement assez court, de l'état d'urgence sanitaire, puisqu'ils ne servent à rien et peuvent constituer un danger sanitaire.

Comme les délais de la rétention administrative ont été protégés- ils peuvent aller jusqu'à trois mois -, il est tout à fait possible de maintenir ces anciens condamnés en centre de rétention administrative dans des conditions

naturellement à toutes les autorités administratives indépendantes qui ont vocation à défendre les droits de l'homme de le vérifier. Quel est

Voilà comment se mettra en place un dispositif qui doit permettre, à partir d'un patient zéro, de remonter toute la filière des contaminations possibles, en dévidant la pelote de laine. Comment voulez-vous faire tout en vous appuyant uniquement sur le médecin de famille ? C'est impossible. Absolument ! Le médecin de famille peut être plus ou moins coopératif- nous souhaiterions évidemment qu'il le soit le plus possible.

la commission des affaires sociales et la commission des lois ont voulu accumuler les garanties. En termes de contrôle, la mise en place d'une instance indépendante chargée d'auditer le fonctionnement de ce système d'information. Ce point est extrêmement important. Nous voulons

Nous sommes capables de le faire- ce n'est pas que cela nous plaise. Nous faisons de notre mieux pour lutter le plus efficacement possible contre ce fléau sanitaire.

le ministre, la volonté du Gouvernement de bien faire dans la recherche de solutions innovantes. Nous sommes tous très conscients qu'il faut trouver les voies et les moyens de combattre efficacement ce virus.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

afin d'identifier leurs proches. Un temps envisagée, l'application mobile StopCovid semble avoir été abandonnée au profit d'un système plus humain de brigades anti-Covid.

Les brigades d'anges gardiens, la terminologie militaire initialement employée ayant été adoucie par un emprunt au vocabulaire religieux, constituées seulement de 5 000 agents de l'assurance maladie, auront pour mission d'informer les personnes susceptibles de porter le virus. Liant fichage des malades, traçage des personnes et recueil des données personnelles et médicales, ce dispositif paraît particulièrement attentatoire au respect de nos vies privées. L'application StopCovid semblait intrusive, les « anges gardiens » des brigades le seront davantage et sans garantie d'efficacité. On se demande si l'exécutif ne navigue pas à vue.

gaz ? Le Premier ministre prétendait récemment vouloir protéger, tester, isoler, mais seule la dimension de l'isolement est présente dans ce projet de loi. Aucune stratégie relative au dépistage massif des Français n'a encore été révélée.

Aussi voudrais-je éviter de brandir immédiatement l'étendard des libertés publiques, même si j'en aurais bien envie, celui de la souveraineté numérique, ou encore celui des quarante ans de combat pour garder ou retrouver la maîtrise de nos données personnelles évoqués

Un système centralisé national agrégeant nos données médicales avec identification est-il indispensable ?

débattre avec vous. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'ouverture de la séance de ce soir pour poursuivre et terminer l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.